Les textes prévoient en effet que les mairies peuvent, de leur propre initiative, instaurer chaque année une taxation sur les locaux commerciaux qui ne sont plus utilisés. Le but est d’inciter les propriétaires soit à relouer leur bien, soit à le vendre. Cependant, cette mesure souffre de plusieurs limites. Tout d’abord, la mise en œuvre de la taxe, bien que décidée par la commune, dépend du service des impôts du département concerné, qui en fait l’examen en fonction des éléments adressés par le propriétaire, et non des éléments factuels relevés par la commune. En ce sens, certains locaux peuvent être vacants depuis plusieurs années ; le cas existe dans la préfecture de la Charente. Dès lors que les propriétaires peuvent démontrer par un quelconque moyen que le bien a vocation à changer de destination, ou bien que celui ci a fait l’objet de travaux, alors ils ne sont pas assujettis à la taxe. Par ailleurs, l’appréciation qui est faite à long terme de ces éléments soulève des interrogations. Certains biens sont vacants depuis plus de dix ans et la taxation n’a pas eu d’effet pour eux. En effet, les propriétaires apportent chaque année un justificatif de travaux minimes, ou une annonce de mise en vente à un prix bien à un prix bien supérieur à celui du marché. Ainsi, la véritable intention de rénover ou de vendre n’est pas contrôlée par les services fiscaux. Quelles actions concrètes le Gouvernement compte t il mettre en œuvre pour exercer un meilleur contrôle, peut être en limitant l’exonération dans le temps,

la lutte contre la vacance commerciale est une priorité majeure pour le Gouvernement. Nous constatons une augmentation inquiétante de cette vacance, tant en centre ville qu’en périphérie, ce qui constitue une véritable préoccupation pour les élus locaux et les acteurs du commerce. Face à cette situation, il est essentiel de repenser l’offre commerciale dans sa globalité. À cet égard, la vacance commerciale fait l’objet d’une « opération nationale 2025 » lancée par les chambres de commerce et d’industrie (CCI), et soutenue par les équipes de la direction générale des entreprises (DGE), afin de mieux mesurer et définir ce phénomène. Parmi les outils à disposition des collectivités pour lutter contre ce fléau figure la taxe sur les friches commerciales (TFC).

le manque de zonage et les conditions d’exonération trop légères freinent son efficacité. Le Gouvernement est conscient de ces difficultés. Une réflexion action

L’analyse de faisabilité est en cours sur les aspects juridiques afin de répondre plus efficacement aux attentes des communes et des acteurs économiques. Je vous assure, encore une fois, que cette question est une priorité pour le Gouvernement. Des mesures concrètes seront proposées dans les mois à venir pour renforcer la lutte contre la vacance commerciale et soutenir la redynamisation des centres villes. Je vous propose, monsieur le sénateur, d’organiser un rendez vous avec la DGE, si vous le souhaitez. La parole

et numérique. Madame la ministre, dans le Calvados comme ailleurs, les élus et les habitants déplorent une atteinte inacceptable aux quatre missions de service public de La Poste que sont le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l’aménagement du territoire et l’accessibilité bancaire. Sur le terrain, bien que la direction de La Poste affirme tout mettre en œuvre pour assurer ces missions, c’est à chaque fois le même scénario diminution des horaires d’ouverture et suppression progressive de certains services et des effectifs, jusqu’à la fermeture définitive du bureau. Dans le même temps est imposé un modèle économique qui fait la part belle au tout numérique et qui ne satisfait personne, d’autant plus qu’il met à l’écart les plus vulnérables. Tout aussi grave, La Banque Postale, censée être le dernier rempart contre l’exclusion bancaire, déserte progressivement nos territoires. Sans parler des distributeurs automatiques de billets (DAB), qui coûteraient trop cher en maintenance et que l’on ferme brusquement… Ainsi, année après année, les fermetures de bureaux de poste pour « absence de rentabilité » se multiplient. Ces bureaux sont remplacés, au mieux, par des agences postales communales (LPAC) ou des relais commerçants (LPRC), qui ne procurent pas le même niveau de services. Dans ce contexte et en responsabilité, les élus – les maires au premier chef soucieux de garantir un égal accès aux services essentiels, n’ont pas d’autre choix que de prendre en charge les dépenses d’investissement comme de fonctionnement de ces « points de contact ». Ils ne sont que trop conscients que, avec la fermeture d’un bureau de poste, c’est tout un écosystème qui est menacé, et avant tout les commerces de proximité, en particulier dans le monde rural déjà fragilisé. Le prochain contrat de présence postale territoriale 2026 2028 devant être signé à la fin de 2025, je souhaiterais connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour stopper l’hémorragie et faire respecter strictement les obligations définies dans la

Dans ce département, le réseau postal demeure significatif avec 189 points de contact, dont 71 bureaux de poste, 81 agences postales communales

concurrent. De manière générale, pour les communes équipées d’un seul DAB porté par La Banque Postale, cet équipement est maintenu et, le cas échéant, renouvelé. Depuis 2021, une dotation annuelle inscrite dans le projet de loi de finances a été mise en place. Les dotations

lieu le 27 mars prochain. Il est encore trop tôt pour annoncer ce qui sera mis en œuvre dans le cadre de ce contrat. Soyez assurée que le Gouvernement est vigilant quant au bon accomplissement par La Poste de ses missions de service public, et que son soutien

mais également des structures d’expertise en aménagement du territoire telles que les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). J’avais déjà posé une question, l’année dernière, sur le risque d’effritement de cette ressource fiscale. fiscale. C’est son recouvrement qui est aujourd’hui en défaut, ce qui remet en cause la viabilité financière de ces services et entités publics. La grande majorité des avis de paiement qui devaient être envoyés aux propriétaires devant s’acquitter de cette taxe ne l’ont pas été depuis plus d’un plus d’un an, presque deux. Selon les estimations, le manque à gagner pour les finances publiques s’élèverait entre 750 millions et 1 milliard d’euros ! Dans un récent communiqué, les services de Bercy nous informent qu’« il y aura effectivement un décalage sur les reversements de taxe d’urbanisme ». Nous apprenons également que, pour les seuls projets d’envergure,

et les associations d’élus locaux. Quels ont été les tenants et les aboutissants de cet échange sur les perspectives de cette taxe ? Au niveau des ressources humaines, le problème demeure entier, avec des formations qui peinent à se tenir et une plateforme «

Ce transfert s’est accompagné du report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement, calée dorénavant sur la réalisation définitive des travaux, ce qui permet d’unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière L’alignement de la taxation en fonction de la réalité des constructions achevées évite ainsi l’émission de taxes pour des projets abandonnés, qui induisait auparavant une annulation de taxation, taxation, insatisfaisante pour les usagers concernés comme pour les collectivités qui devaient reverser les sommes indûment perçues. Un système d’acomptes

Afin d’optimiser les délais de traitement, la liquidation de la taxe d’aménagement s’appuie sur la dématérialisation du processus déclaratif l’outil GMBI, la création la création d’un référentiel des délibérations des collectivités locales et l’automatisation du calcul des taxes d’urbanisme. Cependant, des dysfonctionnements opérationnels ont pu être observés à l’ouverture de ces nouveaux services. du processus déclaratif dématérialisé a en effet pu susciter des interrogations de la part des usagers et aboutir à des erreurs déclaratives qui ont freiné la liquidation des taxes. Les redevables sont toutefois bien identifiés par l’administration et les taxes dues seront, bien sûr, encaissées et reversées aux collectivités. À cette fin, la DGFiP a élaboré un plan d’action pour rendre plus lisible le processus déclaratif. Un parcours digital rénové et accessible est ainsi proposé depuis le 3 février 2025. En parallèle, la DGFiP a sécurisé les éléments déclarés en 2024 pour permettre la taxation de ces dossiers et pour relancer les redevables susceptibles de payer cette taxe qui n’ont pas encore déposé la déclaration attendue. Enfin,

Ce projet d’envergure, symbole de coopération européenne et levier de développement pour la vallée de la Maurienne, permet la création d’emplois et favorise des investissements, notamment grâce au fonds d’accélération des Cependant, au moment de l’accélération des travaux, les collectivités territoriales tirent la sonnette d’alarme, car elles ne perçoivent toujours pas les retombées fiscales légitimement attendues et annoncées de ce chantier.

entreprises (CFE), dont elles sont privées, il serait légitime qu’elles en bénéficient aussi en partie. Malgré une très légère amorce de versement en 2022, de l’ordre d’à peine 2 400 euros pour la seule commune d’Avrieux, aucune nouvelle rentrée fiscale n’a été constatée, et le besoin de ces recettes ne fera que s’accentuer afin d’anticiper le futur d’après chantier du territoire situé autour de la commune de Modane. En dépit de la volonté marquée des entreprises et de Telt de résoudre ce blocage, les collectivités concernées se voient désormais contraintes de refuser la signature de convention avec Telt, seul moyen de se faire entendre, ce qui compromet l’avancement du chantier. Par ailleurs, un réajustement du Fast à la hauteur du montant actuel du chantier sera nécessaire. Madame la ministre, quelles

à la différence entre le montant total de la fraction de TVA affectée au bloc communal et la part fixe. Le Fnaet est réparti de la même manière que la CVAE : au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposables à la CFE, et, pour les deux tiers, des effectifs salariés employés l’année précédente. La part fixe doit consolider les recettes des collectivités et la part variable, soit 208 millions d’euros en 2024, doit les inciter à accueillir de nouvelles activités. Ces règles budgétaires ne permettent pas, dans le droit en vigueur, de reverser ces produits aux communes savoyardes sur le territoire desquelles se trouve le chantier du tunnel euralpin Lyon Turin. Le Gouvernement ne prévoit pas de revenir sur la réforme de la CVAE, dont la compensation une part de TVA garantit des recettes au bloc communal, en particulier aux collectivités hébergeant le chantier Lyon Turin. S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les installations destinées à abriter des personnes ou des biens y sont imposables de fait lorsqu’elles sont assimilables à de véritables constructions qui n’ont pas vocation à être déplacées. Si une entreprise dispose d’un bien soumis à la TFPB pour son activité professionnelle, elle sera redevable d’une CFE établie dans la commune où est situé le bien.

et numérique. Madame la ministre, dans un contexte de recherche d’économies pour faire face au dérapage des déficits publics, je souhaite vous alerter sur un cas de fraude fiscale qui prive la France de recettes importantes. L’entrée en vigueur en 2016 du système d’échange automatique d’informations entre les pays membres de l’OCDE nous a permis de lutter efficacement contre l’évasion fiscale réalisée par l’intermédiaire de comptes bancaires non déclarés détenus à l’étranger.

La principale réside sans doute dans le fait que l’échange automatique d’informations couvre uniquement les avoirs financiers, et non pas les biens immobiliers. La fortune immobilière détenue à l’étranger est donc très majoritairement opaque. En conséquence, nous assistons ces toutes dernières années à une forte croissance des conversions d’avoirs financiers en biens immobiliers détenus à l’étranger, dont l’objectif est d’échapper à ces obligations fiscales.

Madame la ministre, la voix de notre pays compte au sein de l’OCDE. Quelles sont les intentions du Gouvernement pour lutter contre cette technique spécifique d’évasion fiscale qui entraîne un important manque à gagner pour la France ? La parole est

Comme vous l’avez souligné, ces actifs n’entrent pas dans le champ d’application de la norme commune de déclaration (NCD) développée par l’OCDE, qui autorise aujourd’hui l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers entre plus de 120 juridictions. Pour autant, les administrations ne sont pas dénuées de tout pouvoir en la matière. Il est possible d’obtenir des informations immobilières par l’échange de renseignements sur demande pour les États non membres En Europe, la directive du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal permet un tel échange automatique sur des données immobilières entre États membres, à la condition que les administrations fiscales partenaires disposent de telles informations. La situation n’est pas encore satisfaisante. C’est pourquoi le gouvernement français plaide au niveau international pour une extension du champ des normes d’échange automatique d’informations relatives, notamment, aux biens et revenus immobiliers. Cette approche porte ses fruits puisque les ministres des finances du G20 ont donné un mandat clair à l’OCDE aux fins de lancer les travaux et de permettre aux juridictions intéressées d’échanger des informations relatives aux biens immobiliers, en incluant une mention spécifique sur les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entités détenant de tels biens. La France participe aux travaux de l’OCDE en défendant une approche ambitieuse, dont l’objectif est double permettre la plus large participation à ces échanges et améliorer progressivement la qualité des informations échangées. Ces éléments permettront, je l’espère, de vous rassurer sur l’importance que le Gouvernement accorde à ce sujet. La parole

et de l’énergie. Madame la ministre, le Gouvernement a récemment annoncé une modification du cadre de soutien au développement du photovoltaïque en toiture, avec une baisse brutale des tarifs et un recul des objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie Ces décisions suscitent une vive inquiétude au sein de la filière solaire, qu’il s’agisse des entreprises du bâtiment, des exploitants agricoles ou des industriels, qui comptaient sur cette source d’énergie pour réduire leurs coûts et diversifier leurs revenus. En effet, la baisse rétroactive des tarifs risque d’entraîner l’annulation de nombreux projets en cours, alors même que notre pays cherche à renforcer son indépendance énergétique et à répondre à une demande croissante en électricité. De plus, la mise en place d’un mécanisme de dégressivité inadapté pourrait conduire à un moratoire de fait sur les installations photovoltaïques de taille intermédiaire. Nous avons en mémoire le moratoire de 2010, qui avait provoqué la destruction de près de 20 000 emplois dans la filière. Aujourd’hui, les organisations professionnelles alertent sur le risque d’une nouvelle crise et demandent le maintien du cadre tarifaire actuel pour le segment S21, dans l’attente d’un dispositif de soutien mieux adapté aux réalités économiques et industrielles. Dès lors, madame la ministre, quelles garanties le Gouvernement peut il apporter aux acteurs de la filière photovoltaïque pour assurer la pérennité des investissements et des emplois ? Un dialogue avec les professionnels du secteur est il prévu afin de trouver un compromis garantissant la stabilité de cette filière stratégique

L’État soutient depuis de nombreuses années ce secteur. L’arrêté tarifaire dont il est question ici offre un soutien aux installations depuis octobre 2021 et il a été fortement souscrit sur les dernières années, dépassant largement les objectifs qui lui étaient fixés. près de 1 gigawatt de demandes de contrat sur le segment 100 500 kilowatt crête ont été déposées, soit la moitié de la puissance prévue pour l’année entière. Cet emballement nous conduit à ajuster le soutien à ce segment de puissance. De la même manière, pour les petites installations chez les particuliers, l’intérêt est avant tout d’autoconsommer. Lors des dernières années, malgré une baisse de la prime à l’investissement, les demandes de photovoltaïque ont continué à augmenter.

concertation a conduit à faire évoluer le projet d’arrêté tarifaire qui sera publié dans les prochains jours. Dans la continuité de l’arrêté tarifaire, un appel d’offres simplifié permettra d’allouer un volume donné sur le segment 100 500 kilowatt crête, avec un tarif économiquement viable pour les projets. Il sera mis en place dans les prochains mois après des échanges avec la filière.

prochainement publié. Nous poursuivons le dialogue avec la filière pour que le développement du photovoltaïque soit compatible avec les besoins énergétiques du pays. La parole est à M.

Ces projets, bien souvent portés par les collectivités locales, jouent un rôle important dans la transition énergétique, ont des répercussions positives sur la souveraineté énergétique et

et prévisible, afin de préserver la viabilité des projets photovoltaïques, en particulier ceux qui sont portés par les collectivités locales, sans compromettre l’équilibre économique des acteurs impliqués ? Je vous remercie également, madame quelles actions concrètes sont envisagées pour renforcer la concertation avec les collectivités et les acteurs de la filière, afin d’adapter ces évolutions de manière concertée en prenant en compte la diversité des projets en cours et à venir. La parole est à Mme la ministre

modification a été soumis pour consultation au Conseil supérieur de l’énergie le 12 février. Ces discussions, qui ont duré jusqu’à la semaine dernière, ont permis de prendre acte de la nécessité, dans un contexte budgétaire contraint, de différencier le soutien aux grandes et aux petites installations photovoltaïques.

Il était donc nécessaire d’ajuster notre soutien afin d’optimiser tant la production d’électricité que les coûts de raccordement au réseau. Les échanges pour ajuster le décret ont permis d’étudier des solutions. proposé au prochain trimestre est compatible avec le développement de la filière, les acteurs l’ont confirmé. Dans la continuité de l’arrêté tarifaire, un appel d’offres simplifié permettra d’allouer un volume donné au segment 100 500 kilowatts crête, en garantissant un tarif viable économiquement pour les projets. Il sera mis en place dans les prochains mois, après des échanges avec la filière. Les collectivités feront l’objet d’échanges dédiés. Un arrêté permettant le soutien des petits projets photovoltaïques au sol sera également prochainement publié. Vous l’avez compris, le dialogue ne sera jamais rompu avec la filière, pour que le développement du photovoltaïque soit compatible avec les besoins énergétiques du pays. La parole

sociale et solidaire. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des petits commerces, qui font face à une concurrence de plus en plus rude de la part des géants du e commerce, lesquels accentuent leur domination et fragilisent nos commerces de proximité. Pourtant, les commerces de détail sont essentiels à l’attractivité de nos territoires, notamment en zone rurale. Depuis plusieurs années, des propositions ont été formulées pour instaurer une fiscalité plus équitable. Nous avons notamment envisagé la création de taxes sur les livraisons du e commerce ou sur l’artificialisation des sols liée à la construction de grands entrepôts, mais ces propositions sont restées sans suite. Pendant ce temps, la concentration des géants du e commerce s’accélère, avec des conséquences préoccupantes pour nos commerçants, notamment dans les territoires ruraux comme le département de la Manche. Les commerces doivent pouvoir s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et anticiper les évolutions du marché plutôt que de les subir. Or, à la différence de l’artisanat ou du tertiaire, le commerce dispose de peu de dispositifs de soutien à l’innovation. La formation aux compétences numériques doit être renforcée. Nous devons accompagner les commerçants dans la transition vers un modèle hybride, alliant numérique et commerce physique. Certains ont su innover su innover en déployant des systèmes de commande en ligne avec retrait en magasin ou en box sécurisé, mais ces initiatives doivent être encouragées et généralisées. Madame la ministre, les géants du e commerce sont des spécialistes de la logistique avant d’être des commerçants. Il est donc crucial de développer des solutions permettant de les concurrencer sur ce terrain tout en préservant l’interaction humaine qui fait la richesse de nos commerces de proximité. Revoir la fiscalité des grandes plateformes est une piste, mais cela ne peut être la seule réponse. Quelles mesures concrètes le Gouvernement entend il déployer pour accompagner nos commerçants vers le commerce de demain et relever les défis posés au commerce en ruralité ? La parole

L’enjeu majeur est d’accompagner tous les commerçants, notamment les plus petits, dans leur transition numérique. Nous avons par exemple mis en place des dispositifs d’intégration de l’intelligence artificielle. La réunion plénière du Conseil national du commerce prévue en avril prochain favorisera des synergies entre commerçants et start up pour l’innovation. Le Gouvernement soutient également les nouveaux modèles de commerce en zone rurale. Grâce au dispositif national de soutien au commerce rural, il a déjà financé plus de 600 projets pour un total de 14 millions d’euros. En parallèle, le plan de transformation des zones commerciales a été conçu pour porter des projets d’adaptation des zones périphériques. concerne l’équilibre fiscal, les études montrent que la fiscalité des e commerçants et celle des commerces traditionnels sont comparables, les impôts de production représentant 5,5 % de la valeur ajoutée pour les commerces physiques et 5,4 % pour les e commerçants. Il n’y a donc pas de déséquilibre fiscal majeur. surfaces commerciales (Tascom) aux entrepôts logistiques présente des difficultés, notamment en raison de la convergence des modèles physiques et numériques. En outre, une telle mesure risquerait de pénaliser principalement les e commerçants français. Le Gouvernement reste engagé à soutenir l’innovation et à répondre aux défis du commerce de demain à vos côtés, mesdames,

Madame la ministre, depuis plusieurs semaines, l’inquiétude grandit au sujet de la réforme de la procédure d’autorisation des établissements d’accueil de jeunes enfants. Dans le département dont je suis élue, l’Essonne, de nombreux gestionnaires de micro crèches se mobilisent pour sauver leurs structures. déploiement du service public de la petite enfance ne saurait se faire au détriment de ces acteurs majeurs qui offrent des solutions de garde pertinentes pour les parents. Or c’est bien vers une régulation excessive du secteur que l’on se dirige, alors qu’il faut créer 200 000 nouvelles places d’accueil pour répondre aux besoins des familles et que nous manquons dramatiquement de professionnels de la petite enfance. Je ne méconnais pas la nécessité que chaque structure dispose de salariés compétents, possédant une formation avérée en matière de prise en charge du jeune enfant. Nul ne songerait d’ailleurs à confier son enfant à une personne n’ayant aucune expérience en la matière. Mais, de grâce, ne prenez pas des mesures aussi brutales Il est impensable de renforcer la formation des professionnels en poste dans les délais aussi brefs. Je ne suis pas certaine que la date du 1 septembre 2026 fixée pour le recrutement des futurs professionnels qualifiés soit parfaitement adaptée. De même, il me semble incompréhensible que les salariés de nos micro crèches ne puissent évoluer professionnellement au moyen de la validation des acquis de l’expérience si leurs compétences et leurs expériences sont indéniables. Madame la ministre, toute réforme doit faire l’objet d’une concertation approfondie pour être acceptée. Au regard des difficultés du secteur, il est indispensable de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre afin de renforcer la qualité de l’accueil des jeunes enfants et d’améliorer les conditions de travail et de formation des professionnels. Aussi ma question est elle la suivante : le Gouvernement est il prêt à retarder quelque peu cette réforme afin de prendre le temps d’élaborer des solutions pertinentes pour les familles et les salariés et économiquement viables pour les micro crèches ?

Les micro crèches devront compter au moins un professionnel de catégorie 1, et prévoir l’accueil de trois enfants ou moins par professionnel. Par ailleurs, un directeur ne pourra exercer des fonctions de direction que pour deux établissements au maximum. Toutefois, ce décret n’entrera en vigueur qu’à compter du 1 septembre 2026. Les auxiliaires de puériculture ou tout autre professionnel occupant le poste de référent technique avant cette date pourront être maintenus sur leurs postes. Tous les titulaires d’un CAP présents dans les crèches n’auront pas à acquérir le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture et pourront continuer d’exercer. En effet, de nombreuses crèches disposent déjà d’un directeur pour deux structures et comptent 40 % de personnel de catégorie 1.

Enfin, pour reconnaître l’engagement des professionnels et renforcer l’attractivité des métiers, le Gouvernement entend faciliter l’accès au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture ou tout autre diplôme appartenant à la catégorie 1, par voie de

de la protection de l’enfance. Le Gouvernement partage votre position et vos préoccupations : la prévention spécialisée est une mission essentielle pour protéger les enfants. Elle favorise l’insertion des jeunes risquant la marginalisation et contribue à la cohésion sociale. Pour ce faire, des actions éducatives et sociales de proximité sont menées directement auprès des jeunes et de leurs familles.

La jurisprudence a reconnu le caractère obligatoire de ces dépenses lorsqu’il existe sur le territoire du département des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale. Toutefois, les départements peuvent définir les conditions d’exercice de cette compétence selon les Pour mettre fin à la réduction des moyens accordée à la prévention spécialisée, la contractualisation que l’État passera avec les départements en 2025 visera à inciter ces derniers à s’engager pleinement dans ce dispositif. À ce titre, la contractualisation doit s’adapter à de nouveaux enjeux, comme celui de l’utilisation croissante d’internet par les jeunes ou le repérage précoce des souffrances et de la radicalisation. Il existe également un enjeu de formation pour étayer la spécialisation des éducateurs de rue. De son côté, l’État est directement intervenu pour soutenir la prévention spécialisée au travers de différentes politiques publiques. Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, de nombreux clubs de prévention spécialisée ont été lauréats d’appels à projets. dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté, 5 millions d’euros par an ont permis de développer des actions de prévention spécialisée afin d’aller vers les publics qui rencontrent Dans le cadre des politiques de prévention de la délinquance, le fonds interministériel de prévention de la délinquance finance des actions de prévention spécialisée…

Toutefois, la fermeture prévue des deux hôpitaux précités inquiète les soignants, les habitants et les collectivités territoriales. Ces deux sites accueillent en effet plus de 80 000 passages annuels aux urgences et offrent une capacité combinée de plus de 1 000 lits. Depuis

pouvez vous préciser le plan de financement et le calendrier prévu pour l’ensemble du projet d’hôpital Grand Paris Nord ? De plus, pouvez vous nous assurer que les maires des arrondissements et des villes concernées par ce projet seront consultés pour toutes les phases des travaux ? La parole est à Mme la ministre

Le recentrage de l’offre de soins vers la Seine Saint Denis ne déstabilise pas l’offre du nord de la capitale. Le campus nord de Saint Ouen est situé dans la même zone de recrutement que les hôpitaux Bichat et Beaujon, à quelques centaines de mètres du site actuel du premier. L’hôpital de Saint Ouen comportera 986 lits, avec 105 places d’hôpital de jour de plus qu’aujourd’hui, permettant 35 000 hospitalisations de jour supplémentaires par an. Le regroupement des deux établissements, la densification du plateau technique et le renforcement massif des lits de soins critiques permettront quant à eux d’améliorer la fluidité de la prise en charge.

concerne le calendrier des opérations, les travaux de démolition et de dépollution ont été finalisés en avril 2024. L’instruction de la demande d’autorisation environnementale commune du campus est en cours. Pour le site principal, le dépôt des dossiers de demande de permis de construire a été effectué à la mi février 2025. Les consultations et attributions du marché de travaux auront lieu en 2025 et en 2026. Les travaux de construction débuteront quant à eux en janvier 2026 pour s’achever en 2032.

alors qu’un vaste plan de contrôle était lancé dans toutes les régions pour s’assurer de la qualité et de la sécurité des accompagnements proposés aux personnes âgées dépendantes. Le temps a passé depuis, mais tous les professionnels restent inquiets au regard de l’état des finances des établissements – selon

d’euros dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 permette de mieux faire. Il y a deux semaines, la Fédération hospitalière des Hauts de France signalait ainsi que, en raison d’un déficit trop important, une dizaine d’Ehpad publics pourraient être amenés à fermer en 2025, alors même que six Ehpad publics ont déjà fermé dans la région en 2024. À cette situation financière précaire s’ajoute le manque de personnel dédié à la dépendance. Les aides soignants des Ehpad étant financés à 70 par les agences régionales de santé et à 30 % par les départements, il est évident que dans un département peu riche comme le Nord les embauches sont moins faciles. Les premières victimes de ce manque de personnel sont évidemment les personnes âgées elles mêmes, qui sont moins bien accompagnées, voire parfois maltraitées, mais les professionnels souffrent aussi de la dégradation de leurs conditions de travail. Pour toutes ces raisons, au delà des crédits votés pour 2025, pouvez vous nous dire, madame la ministre, quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre afin d’améliorer la situation des Ehpad publics dans notre pays ?

pour personnes âgées dépendantes publics, et en particulier sur celle de l’Ehpad Saint Aile, situé sur le territoire de la commune de Rebais, en Seine et Marne, département très durement touché par les inondations. J’ai été récemment sollicitée par plusieurs élus et habitants du territoire qui ont des parents résidant dans cet établissement. de la situation matérielle, qui a été aggravée par les épisodes orageux et pluvieux de ces derniers mois. Aujourd’hui, comme pour un grand nombre d’établissements de ce type, un investissement important est devenu incontournable pour assurer la pérennité du bâtiment, réparer les dégâts récents et opérer les différents travaux utiles à l’amélioration de l’édifice. Les départements font le maximum pour soutenir ces établissements, mais leurs moyens financiers sont extrêmement contraints. Le conseil départemental de Seine et Marne a déjà accordé à l’Ehpad Saint Aile une subvention exceptionnelle de 300 000 euros en novembre dernier, mais il ne peut aller au delà. Les collectivités locales ne peuvent malheureusement plus porter seules les investissements importants pour la réhabilitation, la rénovation et la reconstruction de ces bâtiments. Un soutien de l’État est indispensable pour les appuyer. Madame la ministre, quelles formes de soutien direct ou indirect envisagez vous en faveur de ces structures ou des collectivités locales qui en ont la responsabilité ?

ont permis de soutenir l’investissement dans le secteur médico social pour des opérations de restructuration, de création, d’extension et de mise aux normes des Ehpad. Les

Dans le cadre du Ségur de la santé, les plans d’aide à l’investissement ont connu un essor important de 2,1 milliards d’euros durant la période 2021 2024,

de l’autonomie et du handicap. Madame la ministre, vingt ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, force est de constater que le handicap est toujours indétrônable sur le podium des discriminations. En démocratie, voter n’est pas seulement un droit, c’est un acte citoyen fondamental. Or, bien que garantie par l’article 29 de la convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, ratifiée par la France en 2010, la participation des personnes en situation de handicap à la vie politique et publique fait face encore aujourd’hui à de nombreux obstacles. Ce constat est partagé par l’Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées (APHPP), entendue en audition au Sénat par le groupe d’études sur le handicap, présidé par ma collègue Marie Pierre Richer, que j’associe à ma question. Certes, des recommandations permettant d’améliorer l’accessibilité des campagnes électorales ont été émises par le Gouvernement, telles que la mise à disposition des documents de campagne en français facile à lire et à comprendre (Falc), mais cela ne suffit pas. Ces bonnes pratiques doivent désormais être rendues obligatoires, avec, par exemple, une phase d’incitation dès les élections municipales de 2026, suivie d’une obligation pour les scrutins ultérieurs. Une étude sur le coût réel de l’accessibilité pourrait également être envisagée pour permettre le déplafonnement des comptes de campagne, afin d’éviter que les candidats ne limitent leurs efforts d’inclusion.

Ainsi, afin que ces personnes ne subissent pas, en plus d’une peine sociale, professionnelle et familiale, une exclusion de la vie citoyenne, pouvez vous nous préciser, madame la ministre, les mesures que vous envisagez de prendre pour garantir, dès les prochaines échéances électorales,

plusieurs mesures ont été adoptées visant à permettre l’accessibilité physique du processus électoral. En amont de l’élection, des consignes précises sont passées aux organisateurs de scrutin en matière d’accessibilité physique des bureaux de vote. Pendant l’élection, le président du bureau de vote doit prendre toute mesure utile pour faciliter le vote autonome des personnes en situation de handicap. Enfin, en aval de l’élection, le ministère de l’intérieur organise des retours d’expérience qui permettent de recueillir tout signalement relatif à un manquement dans l’accessibilité des bureaux de vote. trois autres axes majeurs de progression sont intervenus. Premièrement, les obligations en matière d’accessibilité de la propagande et de la campagne électorales ont été renforcées. Deuxièmement, les démarches électorales en ligne « Interroger sa situation électorale » et « Demander son inscription sur les listes électorales » ont été rendues accessibles

des processus électoraux et, plus largement, l’engagement dans la vie publique des personnes en situation de handicap. C’est pourquoi le ministre de l’intérieur travaille, par exemple, à la rédaction d’un guide de bonnes pratiques à destination des partis et des candidats sur la rédaction de la propagande électorale

Cela permettra d’associer les partis politiques, les associations de représentants et l’administration. Ce sera le lieu adéquat pour échanger sur les différentes mesures que vous évoquez aujourd’hui, afin de progresser.

de l’accès aux soins. Madame la ministre, ma question porte sur le sujet récurrent de la facturation des indemnités kilométriques des infirmiers. Celle ci repose sur deux conditions figurant à l’article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels

une agglomération est l’« espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux » spécifiques. Par conséquent, un infirmier doit pouvoir facturer les indemnités kilométriques si le domicile du patient se trouve au delà des panneaux d’entrée et de sortie de la ville, même si les adresses se situent dans la même commune.

C’est pourquoi des négociations flash avaient été lancées à l’été 2023, à la demande de ses services, afin d’accompagner les professionnels de santé paramédicaux face à l’inflation.

Cette méthode permet aux acteurs de s’accorder en amont sur la notion d’agglomération, afin de mieux répondre à leurs spécificités territoriales. Elle doit permettre d’éviter les contentieux ; l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence que vous mentionniez incite d’ailleurs à cette déclinaison locale de la notion d’agglomération.

à l’ouverture de négociations conventionnelles ; c’est un engagement auquel le ministre est particulièrement attaché. La soins. Madame la ministre, alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale pour garantir une prise en charge renforcée des troubles psychiques, comment pouvez vous justifier le démantèlement du service de psychiatrie de l’hôpital Cochin Tarnier ? Cette décision est contraire à l’engagement affiché par le Gouvernement en faveur de la santé mentale, dans un contexte où les besoins en soins psychiatriques ne cessent de croître.

Une solution, validée par une large majorité des acteurs médicaux, consistait à déménager et à regrouper cette unité au sein de l’ancien bâtiment de la crèche de l’hôpital Cochin. sous couvert de rationalisation économique, il a été décidé de déménager ce service dans un hôpital gériatrique désaffecté, à distance de Cochin, en attendant une hypothétique intégration à l’Hôtel Dieu, en dépit de l’intérêt des malades. Cette décision va nécessairement entraîner une diminution de l’offre de soins, contrairement aux engagements du Gouvernement. Il n’est pas trop tard pour reconsidérer cette décision et ramener cette unité au cœur de ce

L’université Paris Cité et la Ville de Paris portent un projet ambitieux d’institut pour la santé des femmes, qui sera implanté à Tarnier. Pour engager la transformation de ce site, il a été demandé à l’Assistance les espaces dont elle était occupante. Des solutions d’implantation ont été identifiées pour l’ensemble des activités qui s’y tiennent encore. Parmi ces activités figure une unité de psychiatrie assurant une activité ambulatoire, qui a vocation à rejoindre définitivement le site du nouvel Hôtel Dieu après réhabilitation. Entre la libération de Tarnier et l’ouverture de l’Hôtel Dieu, il est donc nécessaire de trouver une implantation provisoire de cette unité, pour environ trois ans. Plusieurs solutions transitoires d’implantation ont été étudiées. La solution retenue est celle d’une implantation temporaire dans les locaux vacants de l’hôpital de la Collégiale, situés à environ un kilomètre de Cochin. La solution d’une implantation dans la crèche de Cochin a été écartée pour deux raisons : un coût de réhabilitation disproportionné par rapport à la durée de l’opération et une durée de travaux incompatible avec le calendrier de la libération de Tarnier, attendue pour l’été prochain. faire en sorte que les meilleures conditions soient réunies, une mission a été confiée à Édouard Couty, président du conseil hospitalier de territoire du groupe hospitalo universitaire de Paris Centre. Cette mission a permis de confirmer que les conditions d’implantation du service concerné dans le futur Hôtel Dieu étaient conformes aux intérêts tant des professionnels que des patients. patients. Elle a également confirmé que les locaux de la Collégiale étaient adaptés pour accueillir l’unité de Tarnier pendant la durée nécessaire à la finalisation des travaux de l’Hôtel Dieu. Par ailleurs, un plan d’action est en cours de mise en œuvre pour renforcer à court terme la psychiatrie de liaison assurée à Cochin. Affaiblir l’offre en psychiatrie au moment où les besoins n’ont jamais été aussi importants serait bien sûr inconcevable. Le renforcement de l’offre de prise en charge en psychiatrie est au cœur de nombreux projets d’envergure de l’AP HP. Comme vous venez de l’indiquer, madame la ministre, c’est inconcevable et pourtant, vous allez le faire… La poursuite de ce déménagement va entraîner la diminution de 75

L’amyotrophie spinale est une maladie génétique rare et grave, qui entraîne une dégénérescence neuromusculaire irréversible. Elle se caractérise, dans sa forme la plus sévère, par une paralysie et un décès prématuré, souvent avant avant l’âge de deux ans. En France, quelque 100 à 200 nourrissons sont diagnostiqués chaque année, ce qui fait de la SMA la maladie génétique la plus fréquente responsable de la mortalité infantile. Des avancées thérapeutiques récentes offrent de nouvelles options pour traiter l’amyotrophie spinale, à condition que le traitement soit administré précocement. En juillet 2024, la Haute Autorité de santé (HAS) a émis un avis favorable sur l’intégration de la SMA dans le programme national de dépistage néonatal. Or, huit mois plus tard, cette recommandation n’a toujours pas été appliquée, mettant en danger la vie de nombreux nourrissons. Un dépistage précoce et une prise en charge rapide offriraient pourtant une chance réelle à ces jeunes enfants. Aussi, madame la ministre, pouvez vous nous indiquer quand le Gouvernement prévoit de mettre en œuvre le dépistage néonatal national

Vous avez raison, le dépistage néonatal constitue un levier essentiel de prévention et de prise en charge précoce des maladies rares. C’est pourquoi le Gouvernement s’est engagé dans une dynamique d’élargissement progressif du programme national de dépistage néonatal, conformément aux recommandations de la HAS. En 2025, trois nouvelles pathologies seront intégrées à ce programme, dont l’amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire grave dont la prise en charge précoce change radicalement l’évolution, comme vous l’avez souligné. Les travaux de mise en œuvre pour ces trois extensions sont bien avancés ; les appels d’offres pour les équipements nécessaires ont été lancés ; les procédures d’agrément en génétique ont été clarifiées, sans obstacle réglementaire ou organisationnel pour les laboratoires des centres régionaux de dépistage néonatal. Par ailleurs, une formation en agrément limité en génétique, pour les quelques professionnels de santé concernés, est en cours de finalisation au sein de l’Agence de la biomédecine. Ces travaux préparatoires sont indispensables, mais ils nécessitent un temps incompressible. Nous essayons néanmoins d’anticiper ce qui peut l’être agences régionales de santé (ARS) de poursuivre très activement les travaux préparatoires. Ainsi, une note d’information demande aux acteurs d’engager dès à présent les préparatifs nécessaires à l’acquisition des équipements et au recrutement du personnel requis. En outre, un arrêté encadrant ces trois extensions fait actuellement l’objet des consultations obligatoires, en vue de sa publication d’ici à la fin du mois mars ou au tout début du mois d’avril. Cet arrêté fixera l’extension du dépistage néonatal à ces trois maladies, selon un calendrier permettant de tenir compte des dernières étapes nécessaires, telles que l’aménagement des nouveaux équipements et la formation des professionnels, pour garantir la réussite de cette extension. Comme vous pouvez le constater, madame la sénatrice, le Gouvernement est pleinement mobilisé et continue de travailler en étroite concertation

aux maladies vectorielles, notamment à la maladie de Lyme. La Haute Autorité de santé a été saisie pour harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire. En février dernier, elle a publié des recommandations fondées sur une analyse scientifique et rigoureuse, issue incluant experts et associations de patients. Ces recommandations aideront les médecins généralistes à traiter les formes simples et prévoient l’orientation des cas complexes vers les centres spécialisés. concerne le syndrome post traitement de la borréliose de Lyme, la HAS décrit les démarches diagnostiques et thérapeutiques adaptées. Elle rappelle qu’aucune preuve d’infection active ne justifie une antibiothérapie prolongée, reste donc non recommandée. La prise en charge doit être personnalisée, globale et pluridisciplinaire, incluant un soutien psychologique et une réadaptation physique. La HAS préconise également une recherche plus importante, vous l’avez dit, sur les mécanismes et sur les traitements efficaces. Les centres de référence, financés par le ministère, ont commencé ces travaux et les poursuivront dans un cadre strict.

Un groupe de travail réunissant experts, chercheurs et représentants de patients a élaboré un programme, avec pour objectif d’améliorer la prise en charge, la prévention et le traitement de ces maladies. La création de deux cohortes de patients permettra d’enrichir nos connaissances.

de la santé et de l’accès aux soins. La musique adoucit les mœurs, dit on, mais on pourrait aisément convenir qu’elle apaise également les corps et les âmes. Au travers de la musicothérapie, de nombreux patients présentant des troubles psychiques ou neurologiques sont régulièrement soignés, grâce à la pratique ou à l’écoute de la musique.

À ce jour, l’Europe compte onze pays où la musicothérapie est reconnue et réglementée, dont le Royaume Uni et l’Allemagne. La France n’a malheureusement pas encore passé ce cap, alors même que cette pratique est déjà intégrée à de nombreuses structures médicales ou médico sociales de notre pays. L’absence d’une réglementation et d’une organisation claire empêche la rationalisation de la profession. En reconnaissant cette pratique médicale, l’État favoriserait une meilleure formation des professionnels ainsi qu’un accès plus équitable des patients à ce type de soin. Alors que le nombre des maladies psychiques croît en France, qu’entendez vous mettre en œuvre, madame la ministre, pour que la musicothérapie soit reconnue comme discipline médicale, permettant ainsi de structurer une profession qui ne demande qu’à l’être ?

Vous souhaitez savoir s’il est possible de reconnaître cette pratique comme discipline médicale. À ce jour, cela n’est pas envisagé. D’abord, il n’est pas démontré que cela nécessiterait des compétences uniquement médicales ; des professions paramédicales ont ainsi ainsi déjà recours à l’emploi de musique et se forment en conséquence pour accompagner la prise en charge de patients. Ensuite, la France est confrontée à une situation de faible démographie médicale. La fin du, que le ministre de la santé appelle de ses vœux, le renforcement des capacités de formation des médecins,

Dans le département des Alpes de Haute Provence, une équipe, formée d’un délégué militaire, d’un délégué militaire adjoint, d’un officier supérieur, d’un sous officier adjoint et d’un secrétaire civil de la défense, s’engage sans relâche pour maintenir le lien entre État et Nation de manière concrète et visible. Au delà du travail auprès des élus et avec nos anciens combattants, ainsi que de l’entraînement d’une réserve opérationnelle, notre département compte ainsi sept classes « défense et citoyenneté Cette activité au service du recrutement, de l’encadrement et de la coordination de futurs réservistes est sans nul doute appelée à se développer prochainement.

postes, redéployé. Cette décision a été prise en concertation avec les directions des ressources humaines des différentes armées et les employeurs interarmées, notamment la zone de défense et de sécurité sud. Dans le cadre d’effectifs contraints, l’objectif est de renforcer les capacités de résilience de l’état major de zone de défense, afin de mieux faire face aux crises potentielles, mais aussi en prévision de la planification des jeux Olympiques d’hiver de 2030, qui impliquent directement les armées. La suppression évoquée s’inscrit aussi dans des redéploiements qui visent à soulager d’autres départements, dans lesquels le délégué militaire départemental cumule déjà trop de responsabilités. L’activité militaire dans le département des Alpes de Haute Provence est moins importante que dans d’autres départements de la zone de défense et

plus d’une dizaine –, qui lui permettent de déléguer certaines de ses missions, y compris en direction de la réserve. J’appelle d’ailleurs votre attention sur le fait que d’autres départements, dans lesquels les armées sont très implantées, n’ont pas d’adjoint actuellement. C’est le cas du Var, où les fonctions d’adjoint du délégué militaire départemental sont assumées

dans d’autres départements. La délégation militaire des Alpes de Haute Provence pourra continuer de s’appuyer sur le délégué militaire départemental en titre, sur un sous officier d’active et sur une dizaine de réservistes. Cette suppression permet une réallocation utile aux missions opérationnelles conduites par les armées. La parole

On [doit] faciliter l’accès à l’asile des femmes afghanes. » Il a raison : depuis 2021 et la mise en place d’un véritable apartheid de genre en Afghanistan par les talibans, de nombreuses Afghanes ont fui leur pays. Parmi elles, des dizaines de militantes des droits humains, engagées pour la paix et l’émancipation de leur peuple, ont été contraintes de prendre la route de l’exil face à la terrible répression du pouvoir en place à Kaboul. Leurs récits sont glaçants. Beaucoup de ces militantes qui ont vécu l’enfer se sont réfugiées temporairement au Pakistan tout en formulant des demandes de visas pour rejoindre notre pays. Elles ont choisi la France, patrie des droits de l’homme, pour être en accord avec leurs engagements, mais aussi parce que notre pays, universaliste, considère toutes les femmes afghanes comme éligibles à l’asile. Désormais, leur situation au Pakistan est intenable. Depuis le début de l’année 2025, les autorités y mènent une opération « zéro Afghan », qui consiste des arrestations arbitraires et en des détentions. Un ultimatum a été donné : ces femmes ont jusqu’au 31 mars prochain, dans moins de deux semaines, pour quitter le pays. J’insiste : il y a urgence ! Pour les militantes afghanes, un renvoi dans leur pays serait synonyme de mise à mort. Nous ne pouvons tolérer cela. Pourtant, leurs demandes de visas sont pour l’instant bloquées, n’aboutissant pas. Elles doivent être traitées en urgence. Madame la ministre, ce gouvernement a le pouvoir de sauver ces femmes : vous pouvez accélérer les processus de demande de visa, en accord avec les déclarations du ministre de l’intérieur.

la France a mis en œuvre spontanément et volontairement, dès 2021, plusieurs dispositifs qui permettent, aujourd’hui encore, à des ressortissantes afghanes de rejoindre notre pays en toute sécurité pour y demander l’asile. dès mai 2021, avant même la chute de Kaboul, la France a évacué 623 ressortissants afghans, agents de droit local et leurs familles. Dans le cadre de l’opération Apagan, lancée le 17 août 2021, notre pays a procédé à des évacuations de grande ampleur, en plus des demandes de réunification familiale qui ont fait l’objet d’une instruction accélérée, permettant l’accueil de près de 14 000 personnes à ce jour. Après la fermeture de notre ambassade en Afghanistan, les ressortissants afghans ont eu la possibilité de s’adresser aux représentations consulaires françaises dans tous les pays tiers, dont le Pakistan, pour solliciter un visa leur permettant de rejoindre la France afin d’y demander l’asile. 2,8 millions de ressortissants afghans se trouvent actuellement au Pakistan selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les autorités pakistanaises ont lancé un premier plan de rapatriement en novembre 2023 visant les ressortissants afghans en situation irrégulière. Notre ambassade sur place et le ministère de l’intérieur se sont immédiatement mobilisés et ont depuis fourni plus de 750 visas au titre de l’asile à des ressortissants afghans, dont 260 à des femmes. Depuis la chute de Kaboul, près d’un millier de ces visas ont été accordés à des femmes afghanes. Les services français continuent d’instruire au maximum de leurs capacités les demandes, très nombreuses. Par ailleurs, la France a pris un engagement fort en décembre 2023 en lançant l’initiative « Avec

depuis la Turquie, et cet objectif est porté à 500 pour l’année 2025. En revanche, les conditions, notamment sécuritaires, au Pakistan ne permettent pas d’y déployer des agents pour réaliser des missions de réinstallation. constater, monsieur le sénateur, que le Gouvernement met tout en œuvre pour répondre aux besoins de protection des femmes afghanes, dans le respect de ses engagements internationaux. La parole est la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le décret d’application relatif à la bonification des trimestres des sapeurs pompiers volontaires. Cette disposition, Cette disposition, introduite au Sénat lors de l’examen de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, vise à apporter une juste reconnaissance à l’engagement citoyen des sapeurs pompiers volontaires. En effet, l’article 24 de cette loi a créé un dispositif permettant aux sapeurs pompiers volontaires, justifiant d’une durée minimale d’engagement, de valider des trimestres de retraite. Ils peuvent ainsi compléter leur carrière professionnelle, au titre de la reconnaissance de leur engagement au service des populations. Ainsi, les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d’État.

fois posée, à moi compris ! Aussi, madame la ministre, pouvez vous nous indiquer la date de parution de ce décret, très attendu par ceux qui risquent leur vie chaque jour au service de nos concitoyens ? concitoyens ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Alain Marc, je vous prie d’excuser l’absence du ministre de l’intérieur, qui m’a chargée de vous répondre. Tout d’abord, je tiens à rappeler l’attachement du Gouvernement au modèle français de sécurité civile, fondé, entre autres, sur la complémentarité des statuts qui le composent, à savoir les sapeurs pompiers professionnels, les sapeurs pompiers volontaires, les militaires et les bénévoles. Environ 200 000 sapeurs pompiers volontaires s’engagent au quotidien pour porter secours à nos concitoyens. Cet engagement est remis en question par la possible qualification en travailleur du sapeur pompier volontaire.

que je sais partagé par le Parlement, lequel a adopté cette mesure de reconnaissance. Comme vous le précisez, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 tend à ce que les sapeurs pompiers volontaires ayant accompli plus de dix ans de service

Le ministère de l’intérieur a repris le dossier. Il est favorable à ce que l’attribution de trimestres soit progressive et que ceux ci viennent s’ajouter à des années complètes de cotisations. La concertation sur ce sujet nécessite du temps : il ne faut pas aboutir de nouveau à une situation insatisfaisante pour nos sapeurs pompiers. C’est notamment du fait de l’insatisfaction de ces derniers que nous sommes amenés à retravailler ce dossier. Les travaux interministériels ont repris pour aboutir à une solution sérieuse, qui permettra de mettre en œuvre cette disposition en suivant l’esprit de la loi : elle visera à renforcer la fidélisation de nos sapeurs pompiers volontaires et à reconnaître leur engagement. Comme vous, le ministre de l’intérieur souhaite que ces travaux aboutissent le plus rapidement possible afin de reconnaître l’engagement de nos sapeurs pompiers volontaires, indispensables à la Nation. Vous pouvez être assuré, monsieur le sénateur, de l’implication sur ce dossier du ministre et de ses services pour y parvenir dans les prochaines semaines. La parole

ministre de la justice. Madame la ministre, ma question porte sur les responsabilités concernant la production et la distribution d’amiante, mais aussi, et surtout, sur le délai d’interdiction de cette fibre tueuse comme matériau de construction ou dans les équipements de protection. En effet, si c’est en 1977 que l’amiante a été reconnu cancérigène par l’Organisation mondiale de la santé, il aura fallu attendre vingt ans, soit 1997, pour que la France l’interdise effectivement. Pourtant, l’amiante représente plus de 120 000 victimes connues et des dizaines de milliers à venir. Ce sont autant d’agonies pour les malades atteints de cancer et une anxiété pour ceux qui n’ont pas encore développé de séquelles à cette exposition. Dans mon département, le Pas de Calais, l’association Chœurs de Fondeurs se bat depuis plus de vingt ans pour que les salariés de l’usine Metaleurop exposés à l’amiante obtiennent réparation et reconnaissance du préjudice d’anxiété alors qu’ils ont déjà eu à subir un licenciement indigne, pour lequel certains sont encore en procès. salariés exposés à l’amiante et au plomb sont encore concernés. Nous nous acheminons vers une transaction là où les victimes attendaient une reconnaissance de responsabilité. Pouvait il en être autrement alors que la justice a prononcé un non lieu dans l’affaire Eternit, considérant que les responsabilités individuelles ne pouvaient pas être établies ?

avait agi comme un lobby pro amiante retardant l’interdiction de cette matière, il n’y a pas eu de condamnations pour les acteurs de ce dernier. Le Gouvernement Gouvernement entend il constituer un pôle d’instruction aux moyens étendus pour faire toute la lumière sur le drame de l’amiante et refermer ainsi cette plaie béante dans l’histoire sanitaire et sociale de notre pays ? La parole est à Mme la ministre

Il partage la légitime préoccupation de voir les procédures judiciaires engagées traitées avec toute l’attention et l’efficacité requises. Depuis 1996, comme vous l’avez indiqué, d’importants moyens ont été mis en œuvre afin de faire le traitement des plaintes déposées par les victimes de l’amiante. Désormais, les dossiers d’exposition à cette fibre sont traités par les pôles spécialisés en matière de santé publique des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille, qui en ont fait une priorité, tant du côté du siège que du parquet. Ces pôles ont vu leurs moyens augmenter de manière constante depuis leur installation en 2003. À la fin du mois de septembre 2024, ils ont eu à connaître de 76 procédures relatives à l’exposition à l’amiante depuis leur création, dont 33 étaient toujours Parallèlement, les moyens d’enquête ont été durablement renforcés. L’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique, principal service d’enquête saisi sur ce contentieux, dispose désormais de dix détachements sur l’ensemble du territoire, qui sont tous en mesure de traiter des procédures relatives à l’exposition à l’amiante. En complément, la gendarmerie nationale a spécialement formé de multiples enquêteurs, titulaires de qualifications spécifiques, au sein atteintes à l’environnement et la santé publique, mais également au sein d’autres unités ou services qui peuvent être saisis par les magistrats afin d’apporter leur expertise aux enquêtes pénales. Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, la mobilisation de l’autorité judiciaire sur ce sujet est entière. Nous ne lâchons rien. La parole

Par ailleurs, depuis 2022, les appels soulevés contre les décisions de ce même tribunal sont du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse, nouvellement créée, alors qu’ils étaient auparavant du ressort de celle de Marseille. Il en résulte, pour les justiciables comme pour les professionnels du droit vauclusiens, un éloignement regrettable des tribunaux administratifs. Cela était déjà le cas en premier ressort, cela l’est d’autant plus en appel désormais. L’obligation pour les justiciables vauclusiens de se rendre à une telle distance de leur département d’origine dans le cadre des procédures de justice administrative constitue une gêne importante. Le droit pour chacun de nos concitoyens d’accéder de manière égale à la justice est fondamental. Une plus grande proximité des habitants de Vaucluse avec les tribunaux administratifs est donc souhaitable. Dès lors, madame la ministre, quelle est la position du Gouvernement sur la possibilité d’un redécoupage

de notre pays. Cette création a remédié à l’absence d’une juridiction d’appel spécifique au territoire de l’Occitanie, le contentieux de cette région étant auparavant éclaté entre les cours administratives d’appel de Bordeaux et de Marseille, deux juridictions dont le niveau d’activité était parmi les plus élevés. À ce titre, la future cour était amenée à devenir le juge d’appel des trois tribunaux administratifs de la région Occitanie, à savoir Toulouse, Nîmes et Montpellier, tant pour des raisons de cohérence d’organisation territoriale que de viabilité de la nouvelle juridiction, dont le volume d’activité devait atteindre une masse critique suffisante. Restait à choisir pour le siège de cette juridiction entre deux options solides : Toulouse ou Montpellier. Sur ce point, ce sont des considérations pratiques et budgétaires qui ont permis de retenir l’Hôtel de Lestang, à Toulouse. Ce site était, en effet, à la fois l’option de loin la moins coûteuse et la seule dont l’état du bâti permettait une ouverture rapide. Le ministre de la justice est conscient que les questions de découpage territorial sont toujours redoutables et les réponses qui peuvent y être apportées ne sont jamais exemptes de reproches. Nous avons tous à l’esprit les critiques et les débats, parfois vifs, qui ont accompagné la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Toutefois, le rapport de nos concitoyens à la justice administrative ne doit pas se limiter à une vision relevant de la proximité géographique.

sont concernés : urbains comme ruraux rencontrent les mêmes difficultés dans leurs différentes démarches avec l’administration. La situation est telle que la Défenseure des droits a choisi d’intervenir en dénonçant « la déshumanisation et l’éloignement des services publics » » : « Il n’est pas possible d’imposer à tout le monde d’avoir un smartphone et une connexion internet. » Elle poursuit avec justesse : « Ce qu’on est en train de demander aux usagers, c’est de s’adapter aux services publics alors que la règle est l’inverse : le service public doit s’adapter aux usagers. elle pointe en particulier les populations en difficulté face à la dématérialisation : « Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes précaires, les personnes étrangères, les détenus et même les jeunes. » Enfin, elle plaide pour des accueils physiques : « On a besoin de voir des personnes quand on est en difficulté. » Aussi, n’est il pas urgent, monsieur le ministre, de mettre un terme à cette dématérialisation à outrance,

aux services publics est une priorité du Gouvernement. Pour être en phase avec les attentes des Français, l’action que nous menons s’articule autour de deux points : des démarches numériques de qualité et un accueil humain de proximité. Parce que le numérique ne répond pas à tous les besoins, comme vous l’avez indiqué dans votre question, pouvoir accéder à un agent public est essentiel. C’est pourquoi le Gouvernement a choisi d’investir dans des substituts au numérique dans le cadre du programme France Services, afin de garantir un accueil de proximité polyvalent. Ainsi, plus de 19 millions

Lorsque cette absence est la conséquence de l’exercice d’un mandat syndical agricole, les agriculteurs bénéficient de cette prestation à un coût réduit, grâce au concours de l’État. Il s’agit d’une aide financière appréciable et qui se justifie par leur engagement syndical et sociétal. En revanche, les nombreux agriculteurs qui s’investissent comme élus locaux, en particulier comme maire, pour faire vivre la démocratie ne peuvent prétendre à aucune aide financière lorsque l’exercice de leur mandat les contraint pourtant à se faire remplacer sur leur exploitation. L’engagement des élus locaux, notamment dans les territoires ruraux et les plus petites communes, est plus que jamais indispensable à notre société. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés n’ont jamais été aussi grandes et la crise des vocations est, hélas ! bien réelle. Aussi, ne pensez vous pas, madame la ministre, que le concours financier de l’État prévu pour les remplacements dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical pourrait être dupliqué

je vous remercie de votre question. Vous soulevez un point important concernant le soutien aux agriculteurs engagés dans la vie locale. Comme vous, je suis consciente de l’engagement essentiel des agriculteurs, notamment des maires, qui contribuent activement à la vitalité

Je comprends parfaitement les enjeux que vous soulevez concernant l’engagement des agriculteurs dans la vie démocratique locale. Comme vous l’avez bien noté, puisque vous souhaitez étendre ce dispositif aux agriculteurs élus locaux,

J’en reviens aux mandats municipaux qui font l’objet de votre question. Les indemnités relatives à l’exercice d’un mandat local, même si je sais que leur niveau est très hétérogène et souvent trop faible – il faut le reconnaître –, doivent permettre de compenser en partie les coûts induits par le recours à un service de remplacement quand aucune autre solution n’a été trouvée. Au demeurant, les questions relatives aux mandats d’élus locaux – vous le savez – ne relèvent pas uniquement de mon champ de compétence. Toutefois, je note votre proposition avec attention tant je souhaite évidemment valoriser le rôle des agriculteurs

de la souveraineté alimentaire. Madame la ministre, je vous interpelle aujourd’hui, car il y a urgence. Comme vous le savez, la progression géographique du loup s’accompagne d’une augmentation des attaques sur les troupeaux. C’est le cas ces dernières semaines dans les Pyrénées Atlantiques. D’année en année, la prédation exercée par le loup s’intensifie, tant sur le plan géographique que numérique, à tel point qu’il n’existe plus véritablement de territoire préservé. Dans les Pyrénées – je le rappelle –, nous avons déjà d’autres prédateurs, notamment l’ours.

Madame la ministre, entre le loup et la brebis, le loup est l’agresseur victime. Il faut reconnaître la violence que représente la prédation pour les éleveurs, passionnés par leur métier, une violence que toutes les indemnisations du monde ne suffiront jamais à compenser. À ce titre, la convention de Berne a approuvé, le 3 décembre dernier, un déclassement du statut de protection du loup, qui passera d’espèce « strictement protégée » à seulement « protégée

Dans ce contexte, mon ministère accompagne financièrement les éleveurs pour protéger leurs troupeaux contre les attaques, grâce à un dispositif arrêté avec les préfets. Celui ci permet de financer le salaire des bergers, les clôtures, les chiens de protection et un accompagnement technique. Ce dispositif permet d’aider plus de 4 000 éleveurs par an, pour un montant de 38,7 millions d’euros en 2024. En complément,

Enfin, vous le savez, nous défendons l’adaptation du statut du loup, qui doit se faire à trois niveaux. Au niveau international, c’est fait : la modification de la convention de Berne est entrée en vigueur le 7 mars. Au niveau

ayant été boycottée par l’ensemble des organisations syndicales, des fédérations de parents d’élèves et des élus, ce qui n’est pas si courant. Ce boycott est le fruit d’une méthode contestée et de renoncements politiques : ceux En effet, seront proposées 180 fermetures de classes dans le premier et le second degrés, avec pour seule justification la baisse démographique, alors que ladite baisse pourrait être – devrait être ! – un levier formidable pour diminuer enfin le nombre d’enfants par classe, comme cela a d’ailleurs été fait par le Gouvernement dans l’éducation prioritaire.

Malgré cette baisse, nous avons fait le choix de conserver les 4 000 postes qui devaient être supprimés – vous le savez. Vous mentionnez le consensus scientifique selon lequel la taille des classes influe significativement sur la réussite des élèves, notamment les plus fragiles. Non seulement nous partageons ce constat, mais nous agissons

pour 100 élèves : l’augmentation est tout de même très significative. Cette hausse du taux d’encadrement se poursuivra à la rentrée prochaine, puisque le nombre moyen d’élèves par classe atteindra un niveau historiquement bas : 21 élèves par classe. À Paris particulièrement, le taux d’encadrement est favorable : 20 élèves par classe en moyenne, soit le deuxième meilleur taux de France métropolitaine, après la Corse. Au regard de la baisse prévue, 160 classes peuvent être fermées sans impact sur le taux d’encadrement. Les retraits d’emplois des rentrées 2023 et 2024 n’ont d’ailleurs pas dégradé le taux d’encadrement, compte tenu de la baisse démographique constatée. Cette évolution nous permet de répondre aux priorités d’une école qui agit pour la réduction de toutes les inégalités, sociales comme territoriales.

Elle a eu lieu, dans le département du Doubs, sous l’autorité du préfet et de l’inspecteur d’académie. Cette instance répond à un triple objectif : favoriser la cohérence des politiques publiques en matière d’aménagement du territoire éducatif ; faciliter les échanges entre l’éducation nationale, les préfectures et les collectivités ; offrir des perspectives partagées quant à l’évolution démographique, au déploiement de l’offre de formation

Le manque de dialogue fragilise les relations de confiance et nuit à l’attractivité des communes rurales, même si le département du Doubs a la chance d’avoir un Dasen de très grande qualité. L’intérêt supérieur de l’élève doit être la boussole du Gouvernement en matière éducative. L’efficacité des observatoires

Dans votre département du Doubs, le nombre moyen d’élèves par classe est de 20,5 : il est significativement inférieur à la moyenne nationale. Les observatoires des dynamiques rurales, que vous mentionnez, ont justement pour vocation de partager avec les élus locaux une vision anticipée, généralement à trois ans, du réseau éducatif en zone rurale. À cet égard, un dialogue étroit existe entre l’éducation nationale, représentée par les Dasen – et je me félicite de ce que vous avez dit sur le Dasen du et les élus locaux, notamment les maires.

Le Gouvernement poursuit donc cette dynamique de renforcement du dialogue entre toutes les parties prenantes, et ce pour le bien être de tous les élèves, qui demeure notre seule et unique boussole. La parole

et de la recherche. Monsieur le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les multiples défis de l’école en Guadeloupe. De multiples facteurs pèsent fortement sur la scolarité et l’insertion professionnelle des jeunes pertes de jours ou d’heures de classe, tensions sociales, problèmes de transport, sensibilité du territoire aux catastrophes majeures, manque d’accès à l’eau dans certains établissements, manque d’enseignants remplaçants et d’assistants d’éducation.

Plus de 1 200 élèves y sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme ou avec des niveaux de formation trop faibles pour leur permettre une insertion sociale. En plus de ces difficultés, l’école en Guadeloupe fait face au défi de l’autorité, avec une recrudescence de débordements et d’actes de violence contre les professeurs. Pourtant, alors que ces défis appellent des moyens humains qui soient à la hauteur de l’enjeu, une nouvelle baisse du nombre d’enseignants est annoncée pour la rentrée 2025 : 22 postes en moins dans le premier degré et 67 postes en moins dans le second degré. La baisse démographique ne saurait être l’unique variable d’ajustement dans des territoires qui souffrent déjà tant. La rectrice de l’académie de Guadeloupe a reçu les représentants des parents d’élèves et les syndicats de personnels pour échanger sur le sujet. Je salue ce dialogue, mais il faudra faire plus

dite continentale. Monsieur le ministre, quelles réponses le Gouvernement entend il apporter aux défis de l’école en Guadeloupe ? Allez vous revenir sur la décision de suppression de postes d’enseignants à la rentrée 2025 ? La parole

L’éducation nationale est pleinement engagée dans la mise en œuvre de politiques éducatives adaptées aux spécificités de l’académie de Guadeloupe, que vous avez rappelées. Pour ce qui est des taux d’encadrement, l’académie enregistre une diminution significative des effectifs dans le premier degré public. À la rentrée 2025, cette baisse se poursuivra, avec une nouvelle diminution de 430 élèves, sans que cela entraîne un moindre encadrement, au contraire, sachant que le nombre d’élèves par classe est déjà passé de 22 en 2017 à 19 à la rentrée 2024. En plus de ce taux d’encadrement exceptionnellement bas, la Guadeloupe bénéficie de dispositifs spécifiques. À cet égard, je rappelle notamment que, depuis 2019, la Guadeloupe est dotée d’un dispositif de soutien scolaire auquel sont éligibles tous les élèves volontaires. Ce dispositif, qui mobilise 420 intervenants, touche 4 000 élèves et a contribué à une nette amélioration amélioration de leurs performances. En outre, l’académie de Guadeloupe a été pionnière, dès 2021, dans le déploiement des contrats locaux d’accompagnement, qui sont aujourd’hui au nombre de 46 et couvrent 40 écoles, 4 collèges et 2 lycées.

de l’ensemble des situations afin de prendre les mesures adaptées. Je précise aussi que la protection fonctionnelle est systématiquement proposée et un accompagnement médico social mis en place. Concernant la mobilité des enseignants dans les îles du sud de la Guadeloupe, des solutions d’hébergement sont mises en place avec les mairies. Par ailleurs, l’académie, en lien avec les collectivités territoriales, sensibilise les autorités organisatrices des transports concernant les effets des horaires des bateaux sur la scolarité des élèves. Je puis donc vous assurer, madame la sénatrice, que le ministère est pleinement engagé

C’est l’un des enjeux, vous le savez, du règlement européen sur la gouvernance des données, applicable depuis septembre 2023. Ce texte vise à créer un cadre juridique facilitant la disponibilité et le partage des données au sein de l’Union européenne.

permettra la création d’espaces de données d’une taille suffisamment importante pour des travaux de recherche scientifique ou d’apprentissage automatique dans des domaines essentiels comme la santé ou la lutte contre le changement climatique.

La jurisprudence est très claire à cet égard ; elle a été précisée tant par le juge administratif que par la Commission d’accès aux documents administratifs. Ainsi doivent être considérées comme activités commerciales non seulement la commercialisation des données elles mêmes, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif. Par conséquent, les collectivités territoriales, saisies d’une demande de communication, disposent de moyens de droit pour s’opposer à une demande qui leur paraît illégitime. Bien plus, en cas de doute, elles peuvent s’appuyer sur les préfectures, qui pourront les éclairer sur le sens de la réponse à apporter à la demande reçue. Concernant le règlement sur la gouvernance des données, il est d’application directe et donc aujourd’hui en vigueur. La loi du 21 mai 2024

Or cette réglementation ne prend pas en compte les spécificités des territoires de montagne, où près d’un logement sur deux n’atteint pas un DPE classé D. Cette situation est principalement due aux failles du mode de calcul du DPE. D’une part, il pénalise les petites surfaces, très nombreuses en montagne, en raison de la méthode de calcul retenue, fondée sur la consommation d’énergie au mètre carré. D’autre part, il défavorise les logements chauffés à l’électricité par rapport à ceux qui le sont au fioul, au gaz ou au bois, alors même que l’électricité, en France, est décarbonée à 92 %. Enfin, il ne tient pas compte de l’altitude et des conditions climatiques spécifiques, qui nécessitent un chauffage plus soutenu. Ces éléments risquent d’avoir des conséquences dramatiques sur le parc locatif en montagne : des logements pourraient massivement sortir du marché dès 2025, ce qui aggraverait le phénomène des « lits froids

Elle reflète donc à la fois le mix actuel et le mix projeté à long terme et s’applique de manière homogène sur tout le territoire. Par ailleurs, plusieurs types de travaux peuvent améliorer significativement la performance énergétique globale d’un logement, même en zone de montagne. Au delà des travaux d’isolation du bâtiment, l’installation d’une pompe à chaleur conduit ainsi à un meilleur DPE que les systèmes gaz, fioul et bois

Ce délai laisse aux propriétaires le temps d’engager les rénovations nécessaires : celles ci sont indispensables pour que la France respecte ses engagements en matière de réduction des consommations d’énergie et d’adaptation au changement climatique. La parole

Ces structures, qui ont été créées par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, exercent depuis plus de quarante ans des missions essentielles de conseil et de sensibilisation, apportant un service neutre et indépendant aux particuliers, aux collectivités et aux professionnels, grâce à des experts en urbanisme, architecture et paysage.

Or la réforme introduite par la loi de finances pour 2021, modifiant le fait générateur de cette taxe, a entraîné des retards significatifs de perception et des risques accrus de non recouvrement, notamment en cas de travaux inachevés ou de non déclaration d’achèvement. Cette situation pénalise fortement les CAUE et affaiblit leur capacité à remplir leurs missions dans nos territoires. Ces difficultés s’inscrivent en outre dans un contexte de faible dynamique de construction et de tensions budgétaires pour les collectivités territoriales, été durement éprouvées par d’autres réformes fiscales. Quelles mesures le Gouvernement entend il prendre pour soutenir financièrement les CAUE, en particulier dans cette période transitoire ? ministre, de rétablir la délivrance de l’autorisation d’urbanisme comme fait générateur de la taxe d’aménagement, afin de garantir des recettes plus stables et d’éviter les risques de non recouvrement ?

n’a donc pas modifié son fait générateur, qui reste fixé à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Les modalités de transfert retenues ont consisté à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d’aménagement de celui des impôts fonciers gérés par la (DGFiP). La date d’exigibilité de la taxe a été décalée à la date d’achèvement des travaux pour faciliter sa liquidation et développer des synergies avec la gestion des impôts fonciers.

est des projets classiques, le report de l’exigibilité de la taxe n’emporte aucun décalage de trésorerie, car l’achèvement des travaux intervient majoritairement en moins de vingt Néanmoins, une modification du cycle de trésorerie peut apparaître pour ce qui est des projets d’ampleur, dont la construction s’étale sur plusieurs années. Dans ce cas, le dispositif d’acomptes mis en place

Dans cette situation, il est prévu que la prime soit versée à l’héritier ou aux héritiers le notaire gérant la succession. Les documents de dévolution successorale, le RIB du notaire et l’attestation de porte fort doivent être fournis et, le cas échéant, la prime doit être versée.

pendant de très nombreux mois – plus de dix mois, dans certains cas –, après transmission des justificatifs sollicités et sans qu’aucune information soit donnée aux ayants droit lorsqu’ils interrogent les services de l’Agence

plus de 2,4 millions de personnes en ont bénéficié afin de réaliser des travaux dans leur logement, pour 11,7 milliards d’euros d’aides publiques ayant engendré 34 milliards d’euros de travaux. Ces chiffres traduisent une montée en puissance rapide du dispositif porté par les ambitions importantes en matière d’économies d’énergie et de lutte contre les certaines demandes, il est vrai, ont pu rencontrer des difficultés pour aboutir dans les délais habituels, mais ces cas restent très limités en comparaison des 540 000 dossiers instruits en moyenne chaque année par l’Anah. Concernant Concernant la situation particulière que vous évoquez des demandeurs décédés ayant bénéficié de l’octroi d’une subvention, elle nécessite un traitement spécifique par les services d’instruction. La subvention étant due à l’héritier, le solde peut lui être reversé par le biais du notaire et sur présentation des justificatifs de qualité d’héritier ainsi que de filiation. Après le paiement de la subvention, la plupart des cas de demandeurs décédés sont signalés à l’Anah quand le paiement n’aboutit pas et est rejeté à la suite de la clôture du compte bancaire associé. Lorsque cette situation se présente, l’Anah met tout en œuvre pour prendre attache avec les héritiers concernés, avec les informations du contact indiqué, pour résoudre la situation et verser l’aide due dans les meilleurs délais, en effectuant l’ensemble des contrôles Au cours de l’année 2024, l’application de cette doctrine a permis de régulariser le versement du solde de la subvention à la suite du décès de l’usager pour 73 dossiers, dossiers, soit 262 580 euros. Il reste aujourd’hui 76 dossiers en cours de traitement dans le cadre de cette procédure. Je vous prie de croire que l’Anah est pleinement mobilisée pour répondre le plus vite possible aux flux des demandes et pour assurer la qualité et la rapidité du traitement des dossiers nécessitant la prise en compte de ces situations individuelles

(DSEC) en élargissant la liste des biens éligibles, d’écarter le principe de reconstruction « à l’identique » ou encore d’étendre les prérogatives du médiateur de l’assurance. Bien sûr, le marché de l’assurance des collectivités est moins rentable que celui des entreprises, mais les collectivités ne sont pas des clientes comme les autres. Elles sont chargées des missions de service public

afin de les accompagner plus efficacement. Dans le département des Alpes Maritimes, comme partout en France, de plus en plus de collectivités rencontrent des difficultés pour accéder à une couverture assurantielle adéquate. Il faut aider aider les maires, madame la ministre ! Leur mandat est déjà marqué par de nombreuses crises. En janvier dernier, dans cet hémicycle, le Gouvernement s’était engagé à proposer des solutions concrètes. Une réforme urgente du système d’assurance des collectivités doit être engagée ! J’interroge donc le Gouvernement sur les nouvelles mesures que vous proposez, car Breil sur Roya – comme vous le savez – n’est pas un cas isolé

travers des dispositifs qui ont fait leurs preuves, tels que le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, qui peut être mobilisé par les collectivités pour financer études, travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels, ou encore la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques. Pour instaurer un climat de confiance entre collectivités territoriales et assureurs, plusieurs actions ont été déjà engagées. En septembre 2023, la conclusion

territoriales. Le BCT a, par ailleurs, pu intervenir, comme c’est le cas pour la commune de Breil sur Roya que vous évoquez à juste titre, madame la sénatrice. La situation n’est cependant pas satisfaisante. S’agissant de l’impossibilité de trouver un contrat, plusieurs propositions ont été émises par la mission d’expertise menée par Alain Chrétien, maire de Vesoul, et Jean Yves Dagès, ancien président de Groupama. Elles rejoignent les conclusions du rapport du sénateur Jean François Husson. Pour répondre à cette situation de déséquilibre, il convient de dynamiser le marché assurantiel, de veiller à la diffusion des bonnes pratiques en matière de commande publique, tout en engageant des mesures à mieux maîtriser la sinistralité. Le Gouvernement travaille actuellement avec les assureurs pour trouver des solutions pertinentes et innovantes. Il faut davantage accompagner les communes afin qu’elles renforcent la connaissance de leur patrimoine et ciblent leurs efforts de prévention, comme l’a fait le maire de Breil sur Roya.

continuent de subir une dégradation de la qualité de leurs services postaux. En Essonne, dans le Calvados et partout dans le pays, nos bureaux de poste ne cessent de connaître un désengagement progressif, quand ils ne ferment pas tout simplement leurs portes. Ce désengagement se traduit très concrètement par des diminutions du nombre d’heures d’ouverture, par la suppression de certains services, par la baisse des effectifs ou par le passage en agence postale communale. Pourtant, conformément à la loi du 2 juillet 1990, La Poste a une obligation légale de maintenir 17 000 points de contact, répartis de façon que 90 de la population se trouve à moins de 5 kilomètres ou de 20 minutes d’un bureau de poste. Au delà des chiffres, quand des services humains de proximité disparaissent, c’est l’âme du service public qui est en jeu. Les postiers, qu’ils soient facteurs ou guichetiers, incarnent bien souvent ce lien social essentiel que le tout numérique ne saurait remplacer, notamment pour nos aînés, ainsi que pour les personnes isolées ou en situation de dépendance. Or, dans nombre de communes rurales, La Poste reste l’un des derniers symboles tangibles de la République. Madame la ministre, le précédent gouvernement avait un temps envisagé une coupe budgétaire de 50 millions d’euros dans le budget alloué à la présence postale pour 2025, heureusement abandonnée depuis. Quelques semaines plus tard, la Cour des comptes a publié un rapport sur la trajectoire financière de La Poste. Celui ci pointe du doigt, non seulement la distribution du courrier six jours sur sept, mais aussi le maintien des 17 000 points de contact sur le territoire. À ce sujet, la Cour des comptes suggère, notamment, des synergies plus fortes avec le programme France Services. Nous craignons légitimement que ces dernières ne soient probablement pas compensées financièrement pour les collectivités. Alors que la désignation du prestataire du service universel postal est attendue d’ici à la fin de 2025, quelle suite le Gouvernement entend il donner aux préconisations de la Cour des comptes, tout en préservant une présence postale réelle, humaine et pérenne ? Pouvez vous nous garantir que le désengagement de La Poste ne se fera pas une nouvelle fois à la charge de nos collectivités ? La parole est à Mme la ministre

La transformation du réseau de La Poste, notamment la diminution des heures d’ouverture et la conversion de bureaux de poste en agences postales communales, suscite des inquiétudes légitimes. je tiens à rappeler que La Poste reste pleinement engagée dans sa mission de service public, avec notamment le service postal universel et l’obligation légale de maintenir 17 000 points de contact, garantissant que 90 % des Français se trouvent à moins de 5 kilomètres ou de 20 minutes d’un bureau de poste. La Poste fait face à des évolutions structurelles majeures, notamment à la chute de 60 % du volume de courrier en quinze ans. Face à ces défis, La Poste adapte son modèle comme elle le peut ; l’État reste attentif à ce que cette adaptation ne se fasse pas au détriment des territoires ruraux.

tout en maintenant une qualité de service. Afin de préserver la présence postale, plusieurs actions sont mises en place. Le développement des agences postales communales et des relais poste en partenariat avec les collectivités permet de maintenir une offre de services de base tout en adaptant les coûts de fonctionnement. L’essor du réseau des 2 800 maisons France Services : 97 % de la population est à moins de 20 minutes d’une maison France Services, où La Poste est un acteur central. Les expérimentations de solutions innovantes, comme les maisons France Services itinérantes, amènent d’ailleurs les services publics au plus près des citoyens les plus isolés. Enfin, La Poste renforce le rôle des facteurs, qui ne se limitent plus

prévoit en effet la réalisation d’aménagements pour rendre la voirie cyclable lors de travaux de réfection d’une voirie en milieu urbain. Le dispositif a été complété par la loi d’orientation des mobilités qui décline une liste d’aménagements possibles. L’objectif de cet article est de profiter des travaux programmés pour réaliser – à moindre coût – la transformation nécessaire de nos villes en vue de l’accueil des cyclistes et de leur circulation de manière sécurisée. Sans méconnaître les difficultés locales qui peuvent se poser, il est nécessaire de conserver cette disposition avec l’ambition qu’elle porte. Pour autant, je ne suis pas opposée à ce que d’autres types d’aménagements, comme les chaussées à voies centrales bidirectionnelles, soient introduits dans le texte dès lors que les conditions de sécurité pour les cyclistes et automobilistes sont remplies. La sécurité de l’ensemble des usagers de la route est une priorité du Gouvernement, soyez en ici assuré. La parole

Il y a quelques mois, a publié un classement des « pires lignes régionales de France ». En deuxième position sur ce triste podium, on retrouve cette ligne Lyon Paray le Monial Moulins sur Allier, dont la pérennité suscite depuis près de dix ans l’inquiétude des usagers et des élus des territoires desservis. Les usagers sont habitués à des retards à répétition, voire à des annulations de trajets. La fréquence des allers retours ne fait que diminuer, réduisant par là même l’attractivité de cette ligne. ligne. Le retrait d’un poste d’aiguillage en gare de Lamure sur Azergues condamne à un cadencement ralenti et à des trajets non croisés qui ne peuvent correspondre aux horaires de travail des usagers se rendant dans la métropole lyonnaise. Pourtant, cette ligne participe au développement de tout un territoire correspondant au desserrement de la grande couronne lyonnaise. Cette ligne historique est aujourd’hui empruntée par de nombreux travailleurs qui alternent télétravail en région bourguignonne et présentiel dans la métropole lyonnaise, ou vice versa.

déjà totalement. Dans un contexte de décarbonation des transports, notamment en milieu rural, pourriez vous nous indiquer clairement les ambitions du Gouvernement pour cette ligne si utile au sud de la Bourgogne, mais aussi à la métropole lyonnaise ? La parole Monsieur le sénateur Fabien Genet, vous m’alertez sur la situation difficile de la ligne TER entre Lyon et Paray le Monial, plus largement sur la question de la desserte ferroviaire des territoires ruraux. L’État s’est engagé aux côtés des régions dans la remise à niveau des petites lignes dans le cadre des volets mobilité 2023 2027 des contrats de plan État région (CPER) : 2,6 milliards d’euros d’investissements sont prévus, dont 780 millions apportés par l’État l’Agence La ligne qui relie Lyon à Paray le Monial nécessite une coordination étroite entre les régions Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhône Alpes concernant l’organisation de l’offre ferroviaire sur l’axe, pour laquelle elles sont pleinement responsables en tant qu’autorités organisatrices. Les travaux à réaliser pour assurer le bon état de la ligne sont, eux, cofinancés par l’État, les régions et SNCF Réseau dans le cadre des CPER : la ligne a déjà fait l’objet d’un investissement significatif de 44 millions d’euros dans le cadre des CPER 2015 2022. Le Gouvernement est particulièrement conscient de l’importance de la desserte des territoires ruraux par les différents modes de transports. Aussi, le volet ferroviaire 2023 2027 du CPER Auvergne Rhône Alpes, en cours de finalisation, prévoit un financement de 10 millions d’euros assuré à 90 % par l’État et SNCF Réseau afin de garantir la continuité des circulations sur la ligne pour les prochaines années.

Alors que nos forêts vont mal et que les maires ont plus que jamais besoin de conseils techniques, de solutions de gestion et d’un accompagnement réglementaire et financier garantissant une gestion plus résiliente et durable,

Après la suppression de 14 postes en 2021, l’ONF s’est lancé en 2023 dans une nouvelle réorganisation avec des suppressions de postes de terrain supplémentaires. Ces réorganisations incessantes mettent à mal toute la filière, les communes forestières, mais aussi les personnels de cet établissement, qui connaît depuis une vague de départs sans précédent. Dans un contexte de crise sanitaire et de changement climatique, et afin de répondre à la demande de proximité des maires, le ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt s’était engagé en novembre 2024 à ce qu’il n’y ait pas de suppressions de postes en 2025.

remercie de me permettre de rappeler l’importance de l’Office national des forêts dans la gestion de nos forêts publiques, ainsi que l’attachement des élus locaux aux missions et moyens du gestionnaire unique des forêts publiques – vous en avez été la porte parole à l’instant.

En revanche, face à des besoins grandissants dans certains secteurs ou sur certaines thématiques, l’établissement peut avoir besoin de redéployer ses effectifs d’une mission à une autre. Ces redéploiements permettent, par exemple, de mieux faire face à l’extension du risque incendie en répondant aux demandes croissantes des élus locaux pour la mission d’intérêt général défense contre les incendies de forêt » ou encore de développer la contractualisation au bénéfice des communes forestières. Dans ce contexte, l’agence ONF du Haut Rhin, dont fait partie l’unité territoriale de la Doller, mène, depuis dix huit mois, un travail associant les personnels afin de répartir les moyens humains au mieux, en tenant compte des enjeux de gestion forestière, dans un département où 80 % des forêts sont communales. Les ajustements de l’organisation projetés se feront à effectif constant pour l’agence ; la réflexion s’appuie sur une analyse de la charge de travail des différentes unités territoriales. Les données des triages de l’unité territoriale de la Doller Basse Largue, montrent notamment une charge de travail globalement supérieure dans les secteurs de montagne de Saint Amarin, Guebwiller, Munster, Kaysersberg ou encore Ribeauvillé par rapport à celle du secteur d’Oberbruck. Les ajustements envisagés pour mieux répartir les personnels sur les différents triages et sur des fonctions transversales stratégiques visent à garantir une présence opérationnelle de qualité, et à renforcer une capacité d’intervention adaptée

cet organisme dans ses missions essentielles.

voire d’agilité, pour mettre en œuvre des solutions concrètes, mais ils sont souvent démunis devant la complexité des démarches administratives ouvrant droit aux financements. J’avais moi même présenté un amendement visant à financer directement les intercommunalités afin qu’elles mettent en œuvre les plans climat énergie. Au passage, je proposais de prévoir une car les 250 millions d’euros votés en 2024 n’étaient visiblement pas suffisants. Or on se retrouve dans le PLF pour 2025 avec seulement 200 millions d’euros. Ce que je souhaite par dessus tout, c’est que vous facilitiez la vie aux collectivités locales pour accéder à ce fonds Il faut en finir avec les usines à gaz d’appel à projets ou à manifestation d’intérêt divers et variés, auxquels personne ne comprend plus rien, et simplifier la vie des élus et de leurs collaborateurs, désespérés devant la lourdeur des procédures. Je suis élu dans l’Aude, département méditerranéen en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Nous sommes confrontés à la fois à des inondations destructrices et à des sécheresses terribles, qui mettent à mal les productions agricoles. Nous n’avons pas de temps à perdre dans des procédures longues et complexes pour accéder à ces fonds pour nous vitaux

en raison de leur rôle clé dans la transition écologique, les collectivités territoriales sont les principales bénéficiaires du fonds vert. En 2024, le programme a bénéficié à plus de 6 245 demandeurs distincts, dont 5 316 sont des communes – 160 d’entre elles se situent dans votre département de l’Aude. En 2025, pour simplifier l’articulation entre les aides, j’ai souhaité, avec le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen, que les règles d’emploi soient décrites dans une circulaire conjointe

Celle ci a été publiée le 28 février 2025, soit quelques jours après l’adoption définitive du budget et sa promulgation. Elle priorise le soutien à l’investissement local en faveur de la transition écologique, en particulier en matière d’adaptation au changement climatique suivant les objectifs du plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc), que j’ai présenté la semaine dernière. En 2025, malgré une baisse de l’enveloppe du fonds vert par rapport à 2024,

hors appel à projets, comme je m’y étais également engagée, et donc sans contrôle des projets des PCAET dès lors que ces derniers sont votés. Les modalités d’accès à cette ressource sont déjà spécifiées par la circulaire du 28 février et les crédits seront bientôt délégués aux préfets de région. Les collectivités ayant adopté un PCAET au 1 mars 2025 bénéficieront de ces crédits, en concertation avec les préfets. Cette nouvelle mesure témoigne de ma volonté de construire un pacte de confiance avec les collectivités territoriales. Mon objectif est qu’elles puissent mettre en œuvre rapidement et facilement leur PCAET afin d’accompagner leur transition écologique, en cohérence avec la planification écologique que je défends au niveau national. La parole est à M.

pour non respect, selon elle, de la directive Oiseaux, du fait de la pratique dans cinq départements du Sud Ouest de la chasse traditionnelle de la palombe au filet. La procédure ayant commencé en 2019, ses arguments sont connus depuis longtemps. Ils sont cependant entachés d’inexactitudes, que ce soit, par exemple, dans la dimension évoquée des pantières ou dans l’affirmation que ces pantières contribueraient au déclin de la tourterelle des bois, qui a déjà intégré le Maroc au mois d’octobre. Par ailleurs, cette chasse est bien sélective en raison de la maille des filets, le déclenchement manuel des pantes et pantières intervenant après une phase d’observation. En outre, loin d’être menacée, la palombe est en pleine expansion, et désormais classée comme espèce nuisible dans plusieurs pays européens et départements français. Vous comprendrez ainsi la colère que l’annonce du 12 février provoque chez les chasseurs du Sud Ouest, qui s’estiment inécoutés et insuffisamment défendus. Il serait malheureux que, dans un tel contexte de défiance, les chasseurs se démobilisent alors que leurs actions pour réguler le grand gibier ou pour le suivi sanitaire des zoonoses dans la faune sauvage sont sont essentielles. Madame la ministre, êtes vous prête à transmettre aux parlementaires les éléments du dossier de défense présentés à la Commission européenne dans le cadre des échanges engagés depuis 2019 ? De plus, êtes vous prête à rencontrer en personne les fédérations

et pour nos territoires du Sud Ouest. Comme vous l’avez rappelé avec beaucoup de justesse, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, estimant que la France ne respecte pas la directive Oiseaux en autorisant la chasse à la palombe au filet dans cinq départements du Sud Ouest. face à cela, je vais avancer les arguments pour prouver, comme vous le dites, que cette chasse traditionnelle très pratiquée dans le Sud Ouest, et jamais remise en cause sur le plan national, doit perdurer. Car vous avez raison, madame la sénatrice : cette décision concerne non pas une espèce menacée, mais le pigeon ramier, une espèce qui est abondante et parfois nuisible, notamment du fait des dégâts agricoles qu’elle occasionne. Ce n’est d’ailleurs pas un sujet de préoccupation pour les associations environnementales, qui préfèrent concentrer leurs travaux sur les espèces menacées de disparition. Je vous rejoins également sur le fait que cette méthode présente des avantages environnementaux au delà de tous les aspects patrimoniaux que vous avez rappelés. Elle est en effet sélective, comme l’ont montré les expérimentations de cet automne, et les captures accidentelles peuvent être relâchées vivantes, ce qui, évidemment, n’arrive pas avec la chasse au fusil. De plus, cette technique n’occasionne pas de résidus et ne perturbe pas les autres espèces. Je vais évidemment associer les chasseurs à cette démarche. C’est ainsi que j’ai pris contact avec la Fédération nationale des chasseurs (FNC) pour nous mettre en ordre de bataille. Je souhaite travailler main dans la main avec les chasseurs, les agences de l’État et les associations pour démontrer que cette chasse est sélective, contrairement à ce que lui reproche la Commission. J’ajoute que ma porte est grande ouverte à tous les parlementaires qui travaillent sur ce sujet pour consolider notre dossier en défense. Je défendrai avec force cette pratique en cohérence avec les différentes notes transmises à la Commission depuis 2019, date de la première mise en demeure de la France sur le sujet. Vous pouvez donc compter sur moi, madame la sénatrice, pour défendre cette tradition qui, je le sais, rassemble les générations. Ancrée dans l’histoire de votre région, elle fait partie de son identité locale et elle célèbre le lien entre l’homme et la nature. C’est aussi cela que je veux mettre en avant. La parole est à M. Hervé Gillé,

Ma question portera non pas sur le financement à proprement parler des dispositifs de rénovation énergétique, mais sur les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales, en particulier par les syndicats intercommunaux, dans la mise en œuvre desdits dispositifs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rénovation énergétique ne s’est pas accompagnée d’une simplification. Bien au contraire, les outils se sont multipliés – Mon Accompagnateur Rénov’, MaPrimeRénov’, MaPrimeAdapt’ créant parfois un sentiment de désordre dans l’organisation des politiques de l’habitat, au détriment, finalement, de l’efficacité et de la qualité de l’accompagnement de l’usager. Plus problématique encore, la création de ces différents dispositifs a mis sur un pied d’égalité des opérateurs publics Gironde, le syndicat interterritorial pour la maîtrise de l’énergie et de l’habitat (Siphem) et des opérateurs privés aux pratiques parfois peu scrupuleuses. Ce mélange des genres peut nuire à la réussite des projets de rénovation énergétique. L’accompagnement est devenu un véritable parcours du combattant, combattant, provoquant même des renoncements. Ce n’est pas acceptable. Ainsi, face à une demande croissante de la part des ménages, il semble nécessaire de renforcer le rôle des opérateurs publics locaux et de rétablir une concurrence équitable. Ma question est donc la suivante : madame la ministre, face aux demandes croissantes ou insatisfaites, quelles solutions envisagez vous pour éviter toute insuffisance des enveloppes financières consacrées aux syndicats intercommunaux et, ainsi, garantir la continuité de l’accompagnement des ménages tout au long de l’année ? La parole est à Mme la ministre.

de votre question, qui permet de mettre en évidence l’importance du service public de rénovation de l’habitat, France Rénov’, et des guichets qui le portent, tel le syndicat interterritorial pour la maîtrise de l’énergie et de l’habitat, en Gironde. Grâce au service public France Rénov’, les Français bénéficient d’un tiers de confiance auprès de qui recueillir une information et des conseils indépendants et faire remonter toute difficulté rencontrée dans un projet de rénovation. L’État est au rendez vous pour poursuivre la consolidation de France Rénov’ à travers les pactes territoriaux qu’il cofinance avec les collectivités. Comme vous le savez, Mon Accompagnateur Rénov’ est l’acteur clé dans le parcours du ménage lorsque celui ci se lance dans une rénovation d’ampleur et souhaite bénéficier de l’aide financière importante de MaPrimeRénov’. Il appuie le ménage du début à la fin de son projet, dans ses aspects tant techniques qu’administratifs. Nous bénéficions d’une année de recul sur le fonctionnement de ce nouvel acteur. Ce dispositif fonctionne bien et s’ancre de plus en plus dans les territoires. Des partenariats vertueux sont noués avec les collectivités, dont nous souhaitons qu’ils se poursuivent

le Proche Orient (UNRWA) qui permet de mener des actions vitales auprès de cette population palestinienne. La France a récemment annoncé attribuer 20 millions d’euros au budget de programme de l’UNRWA. Il s’agit d’une contribution bienvenue et appréciée qui mérite d’être poursuivie. Malgré l’entrée en vigueur des lois votées par la Knesset et les graves décisions israéliennes, l’UNRWA demeure un acteur humanitaire de premier ordre dans un contexte où la suspension de l’aide américaine nuit gravement au financement de ses actions. Devant le Conseil de sécurité de l’ONU, ce 28 janvier, son commissaire général a appelé les États membres à veiller à ce qu’une crise financière ne mette pas brutalement fin aux activités vitales de l’UNRWA. Le budget de programme, soit un des deux fonds de l’UNRWA, le second étant dévolu aux opérations d’urgence, est alloué au fonctionnement général des services dont dépend sa pérennité. Il finance les actions de développement telles que la santé, les services sociaux et l’éducation pour un demi million de filles et de garçons au Proche Orient, ainsi que les salaires des employés de l’UNRWA.

en Cisjordanie, à Jérusalem Est et à Gaza, et dans les pays qui les accueillent – Liban, Jordanie et Syrie. L’UNRWA est en première ligne pour porter secours à la population civile de Gaza. Elle l’est toujours depuis l’entrée en vigueur du cessez le feu, que nous avons appelé et soutenu. Nous rendons hommage aux travailleurs humanitaires et aux personnels de l’UNRWA décédés dans l’exercice de leurs fonctions. Le soutien de la France est notamment financier. Ces deux dernières années, nous avons ainsi soutenu l’UNRWA à hauteur de 96 millions d’euros. Lors de la conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza, au Caire le 2 décembre dernier, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean Noël Barrot, a annoncé une nouvelle contribution de 50 millions d’euros pour la population de Gaza en 2025, dont 20 millions d’euros pour l’UNRWA. Face à l’urgence, le ministre a annoncé vouloir que cette contribution puisse être décaissée dans les meilleurs délais. Ces 20 millions d’euros permettront à l’UNRWA de continuer à fonctionner. La France continue de suivre les efforts de réforme de l’UNRWA. Ils doivent se poursuivre par la mise en œuvre complète et effective des recommandations du rapport indépendant coordonné par Catherine Colonna. Cette réforme doit garantir le respect de la neutralité du personnel, des manuels scolaires et des installations de l’UNRWA, laquelle est indispensable et exigible de tout acteur humanitaire. Nous resterons naturellement vigilants sur ce point. La législation israélienne visant l’UNRWA est entrée en vigueur le 30 janvier dernier. En lien avec nos partenaires, nous avons demandé à Israël de préserver l’action indispensable de l’Office et de respecter ses obligations internationales. Nous l’avons appelé à coopérer avec ses partenaires internationaux, en premier lieu les Nations unies, afin d’assurer la continuité des opérations humanitaires et de garantir l’acheminement massif, rapide, sûr et sans entrave de l’aide humanitaire, ainsi que la fourniture des biens et services essentiels à la population civile.

Des dizaines de milliers de femmes ont manifesté partout en France pour leurs droits. En tête des revendications, on retrouvait la lutte contre les inégalités salariales persistantes entre les hommes et les femmes. Selon l’Insee, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5 % à celui des hommes dans le secteur privé en 2022 et de 22,2 % en 2023. Certes, l’usage du temps partiel a un impact sur ces résultats, mais, si l’on compare les situations à temps de travail égal, l’écart est tout de même de 14,2 %. Ainsi, sur toute une vie, une femme gagnerait 300 000 euros de moins qu’un homme et même jusqu’à 450 000 euros pour les profils les plus diplômés. Cette inégalité se retrouve également dans les pensions de retraite, qui sont souvent bien inférieures pour les femmes. Si l’on continue à ce rythme, selon une experte citée dans le journal du 3 mars dernier, l’égalité salariale ne sera pas atteinte avant au moins l’an 2100. Vous en conviendrez, madame la ministre, ce n’est absolument pas supportable. Ainsi, sur cette question majeure, il faut une politique volontariste et ambitieuse. D’ailleurs, la Cour des comptes elle même a estimé dans un rapport publié en janvier 2025

Ma question est donc simple : quelles mesures concrètes et rapides le Gouvernement compte t il prendre pour corriger enfin les inégalités de salaire et, surtout, cette injustice criante ? La parole

En 2025, dans notre pays, il n’est pas acceptable que des différences de salaire existent encore au détriment des femmes et qu’une part demeure toujours inexpliquée différences de rémunération à temps de travail identique, c’est 14 % de trop. Pareillement, 4 % d’écart à poste comparable ou équivalent, c’est 4 % de trop. L’égalité salariale n’est pas un objectif ; elle figure d’ailleurs dans la loi depuis 1972. En 2019, la France a été le premier pays européen à créer un index d’égalité salariale, car on ne peut corriger ce qu’on ne mesure pas. Depuis lors, 857 entreprises ont été mises en demeure et plusieurs dizaines ont été sanctionnées, jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires, pour non respect de leur obligation de transparence. Nous voulons aller plus loin. Un travail est en cours sous l’autorité d’Astrid Panosyan Bouvet, ministre chargée du travail et de l’emploi, pour transposer la directive européenne de transparence salariale du 10 mai 2023. Elle devra l’être en droit interne d’ici au 7 juin 2026. renforcera les exigences qui pèsent sur les entreprises en prévoyant un droit à la transparence des rémunérations avant l’embauche, une obligation de transparence à l’égard des employeurs relative à la mise à disposition des critères utilisés pour déterminer les rémunérations, les niveaux de rémunération et la progression des rémunérations, une obligation pour les employeurs de fournir, entre autres, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Mais se battre pour l’égalité salariale, c’est aussi, dès le plus jeune âge, permettre à de petites filles et de petits garçons d’embrasser pleinement les carrières qu’ils souhaitent. Cela passe par une action renforcée en faveur de la mixité dans les filières, en particulier celles qui forment à des métiers stratégiques pour notre souveraineté. Cela passe par l’école dès le plus jeune âge, afin de lutter contre les inégalités, d’empêcher que l’on enferme encore trop rapidement les petites filles et petits garçons dans des destins préconçus nourris par la reproduction des stéréotypes. Il est primordial que la lutte contre ces stéréotypes devienne notre priorité absolue.